L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons tous été bouleversés par les drames qu’a connus notre pays, drames causés par des conducteurs en excès de vitesse, sous alcool ou sous stupéfiants.

nourrit l’ambition de répondre à ces critiques. Il est en effet de notre devoir de nous assurer que notre droit prenne pleinement en compte toutes les situations. Il est de notre devoir que notre droit s’adapte aux nouveaux comportements, qui transforment nos routes en voies périlleuses. Il est aussi de notre devoir que notre droit n’aggrave pas, par ses mots, la souffrance des victimes. C’est pourquoi la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui n’est pas que symbolique. Elle propose de nommer juridiquement, avec justesse, des comportements inacceptables, qui favorisent la survenance de drames sur nos routes. Cette proposition de loi n’est pas qu’une œuvre sémantique. Bien évidemment, les mots ont un sens. Mais, en droit, les mots emportent des conséquences sur le déroulement des enquêtes, sur les audiences, sur la prise en charge des victimes. Les mots consacrés par la loi obligent la justice. La qualification pénale d’homicide ou de blessures involontaires n’est pas appropriée lorsque le conducteur s’est délibérément mis dans un état ou une situation faisant encourir un risque avéré aux usagers de la route. L’acte n’est pas totalement accidentel lorsqu’une personne conduit sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Il n’y a rien d’involontaire Il n’y a rien d’involontaire à consommer des stupéfiants ou à s’enivrer. Il n’y a rien d’involontaire à prendre la fuite après avoir commis un accident. À travers le nouveau qualificatif consacré par cette proposition de loi, le caractère inacceptable du délit est ainsi pris en compte. ce texte accroît la répression. De nombreuses mesures visent à renforcer les sanctions en matière routière. Au demeurant, cette proposition de loi s’inscrit dans le prolongement par le Gouvernement le 17 juillet 2023, à l’occasion du comité interministériel de la sécurité routière. Il est vrai que la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière avait déjà consacré des textes d’incriminations spécifiques. À ce titre, l’article 221 6 1 de notre code pénal dispose que « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité […] est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende si l’homicide a été commis avec au moins deux circonstances aggravantes. L’article 1 de la proposition de loi a été profondément remanié par la commission des lois de votre assemblée. Si je salue la créativité et l’inventivité ça comme ça ! … je ne suis pas favorable à la nouvelle architecture qui en résulte. Vous proposez de consacrer une nouvelle forme d’atteinte aux personnes, dès lors qu’elle est causée par un auteur qui n’est pas un conducteur. Ainsi seraient créés un délit d’homicide par mise en danger et un délit de blessures par mise en danger. C’est génial ! Ces deux délits s’ajouteraient alors non seulement aux délits d’homicide et de blessures involontaires, mais également aux délits d’homicide routier et de blessures routières. Pourquoi faire simple, quand on peut faire très compliqué… et de lisibilité de la loi pénale. Exactement ! Lorsqu’une victime est décédée, lorsqu’une victime est blessée, la mise en danger est avérée, indépendamment de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Au demeurant, l’article 1 de la proposition de loi, dans la rédaction emporterait une complexification de notre droit. En effet, coexisteraient alors : une section 1 relative aux atteintes volontaires à la vie la vie ; une section 2 relative aux atteintes involontaires à la vie ; une section 2 relative aux atteintes à la vie par mise en danger ; une section 2 relative à l’homicide routier

L’équilibre actuel de notre code pénal en serait à l’évidence fragilisé. À cet écueil, s’ajoute l’édification d’une frontière dangereusement poreuse entre les infractions non intentionnelles et les infractions volontaires. La qualification de l’infraction soumise aux magistrats deviendrait trop complexe. l’exigence constitutionnelle de clarté de l’incrimination pénale ne me semble pas respectée. Pour toutes ces raisons, je suis favorable au rétablissement de l’article 1, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale. Serait ainsi créé dans le code pénal un chapitre intitulé « Des homicides et blessures routiers », dans lequel seront introduits quatre nouveaux articles. L’homicide involontaire et les blessures involontaires par conducteur, dès lors qu’ils sont aggravés, seraient désormais caractérisés comme étant un homicide routier ou des blessures routières. Les circonstances aggravantes, déjà prévues par le code pénal, D’autres circonstances aggravantes méritent cependant d’être ajoutées, car elles traduisent des comportements malheureusement trop fréquents de la part des conducteurs ; car elles font désormais partie intégrante du quotidien des enquêteurs, des magistrats et des victimes ; car il nous faut être en prise directe avec la réalité, avec le quotidien de nos routes. Le conducteur téléphonant au volant, celui qui se livre à un rodéo urbain et qui provoque la mort d’un usager de la route doit être poursuivi pour homicide routier ou blessures routières. Celui qui consomme du protoxyde d’azote, celui qui suit un traitement médicamenteux interdisant toute conduite, ceux là mêmes qui prennent malgré tout le volant et qui blessent ou tuent, ceux là mêmes doivent être poursuivis pour homicide routier ou blessures routières. Les peines principales encourues pour les faits d’homicide routier ou de blessures routières restent identiques à celles qui sont actuellement prévues pour homicide ou blessures involontaires aggravés. Concernant la répression de l’homicide routier, un amendement du rapporteur en commission à rétablir l’article 132 19 1 du code pénal relatif aux peines planchers – les bonnes vieilles peines planchers Vous le savez, je suis totalement défavorable à un tel rétablissement. Premièrement, les peines planchers n’ont pas démontré leur efficacité.

à 37 % en 2011, les tribunaux ayant dérogé aux peines planchers, qui leur apparaissaient manifestement disproportionnées. Troisièmement, les peines planchers n’ont eu aucun effet sur le nombre de peines d’emprisonnement prononcées et sur leur quantum. Durant les années d’application des peines planchers, soit entre 2008 et 2013, le quantum moyen de la peine d’emprisonnement ferme était de sept mois. Dès l’abrogation des peines planchers, entre 2014 et 2019, le quantum moyen était de huit mois. En 2022, il était de dix mois. Enfin, le rétablissement de peines planchers va aggraver les délais de traitement des dossiers en matière pénale. En effet, ce dispositif suppose un temps d’audience prolongé, afin que le ministère public et les parties échangent leurs arguments sur l’application, ou non, de la peine plancher, et un temps de motivation supplémentaire pour le juge. Je le dis sans polémique, mais de manière claire : je préfère l’efficacité à la démagogie, et je sais que le Sénat aussi ! Je souscris à une répression ferme, fondée sur des peines principales et des peines complémentaires efficaces, prévenant toute réitération. À ce titre, la proposition de loi prévoit d’insérer un nouvel article 221 21 comprenant des peines complémentaires encourues ou obligatoires en cas de condamnation pour homicide routier et blessures routières. En particulier, il est prévu d’élargir la peine complémentaire de confiscation et d’immobilisation du véhicule ayant servi à la commission de l’infraction. Le véhicule conduit, qu’il soit ou non la propriété du conducteur ayant causé le drame, pourra être saisi, puis confisqué. En outre, les dispositions actuellement applicables en matière d’annulation du permis de conduire de plein droit sont étendues à toute condamnation pour homicide routier ou blessure routière ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. De telles propositions visent un objectif louable. Elles permettent de nommer et d’acter la gravité de certains comportements qui sont à l’origine, hélas ! de nombreux accidents. Afin de lutter davantage contre les comportements dangereux au volant et de renforcer la répression à l’égard des auteurs d’infractions routières, le texte répond à ces deux objectifs : l’excès de vitesse de 50 kilomètres par heure devient un délit les règles en matière de récidive sont renforcées ; les peines d’emprisonnement encourues pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants sont aggravées. En conclusion, la loi doit responsabiliser, donc réprimer les auteurs de comportements volontairement dangereux. La loi doit répondre aux évolutions de notre délinquance routière le protoxyde d’azote et de nombreuses substances psychoactives sont trop régulièrement consommés par des conducteurs. En conséquence, la loi doit nommer avec précision de tels délits. L’homicide routier ou les blessures routières sont ainsi les qualifications appropriées dans le cas d’accidents provoqués par le conducteur d’un véhicule ayant commis une faute grave. Il y va tout simplement

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous ne parlons pas de quelque chose d’anodin. Le nombre de morts sur les routes – 3 267 en 2022 – montre qu’il s’agit d’un sujet grave.

une meilleure acceptation sociale d’une telle qualification ». Je ne conteste pas que la loi puisse avoir une portée symbolique.

de ce traitement judiciaire, il m’est apparu choquant que nous divisions les familles en deux catégories : celles qui auraient perdu leur enfant, leurs proches, leur famille

d’accord ! Les auteurs de la proposition de loi ont voulu mettre en avant le caractère délibéré des comportements qui ont permis ce drame.

par heure. Mais nous avons souhaité aller plus loin. La mise en danger de la personne d’autrui n’est pas une invention. Indépendamment de tout dommage, elle a été prise en compte au sein de l’article 121 3 du code pénal dès 1994. En 1996, le manquement aux obligations de sécurité constituait déjà une infraction. En 2000, le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité a même été considéré comme susceptible de constituer un délit, voire un crime. Dès lors, la la commission a voulu inscrire dans le code pénal deux notions qui marquent l’aboutissement de la prise en compte des manquements de l’auteur de l’infraction non intentionnelle les atteintes à la vie par mise en danger ; et les atteintes à l’intégrité physique ou psychique des personnes mises en danger. Ces infractions font apparaître le manquement délibéré à l’obligation de prudence comme une catégorie particulière d’homicide ou d’atteinte à la personne. Elles demeurent néanmoins non intentionnelles et délictuelles, ce qui nous amène au problème des peines. Contrairement à ce que vous pensez, monsieur le garde des sceaux, je n’ai pas la nostalgie de la période que vous avez évoquée. Je ne suis pas animé

à partir de là que le juge doit se poser la question de la détention. Je rappelle que la moyenne des peines dans ce type d’affaires est de seize mois. La peine minimale

Je passe rapidement sur les autres articles du texte qui ont été ajoutés par la commission des lois de l’Assemblée nationale et qui tendent à réprimer davantage la conduite sans permis. La loi,

Havet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous entamons l’examen concerne un sujet extrêmement grave, qui affecte chaque année des milliers de nos concitoyens. Elle traite des violences routières et vise précisément à lutter contre ce fléau. Les chiffres sont alarmants. En 2023, pas moins de 3 402 personnes ont perdu la vie sur nos routes, et rien qu’en février 2024, quelque 224 tragédies supplémentaires sont venues s’ajouter à ce bilan déjà sinistre. La route ne se contente pas de prendre des vies, elle en brise aussi de façon irrémédiable. Il en va ainsi de celles des 232 000 blessés, dont 16 000 graves, recensés rien qu’en 2023. Il est nécessaire de rappeler que, à ces chiffres, correspondent autant de familles déchirées et de destins brisés. Il faut aussi souligner que, aux souffrances des victimes, s’ajoutent l’effroi, la douleur et la sidération qui marquent leurs proches. À leur peine, viennent s’ajouter l’incompréhension et le sentiment amer d’injustice quand on range ces drames sous la qualification d’homicides involontaires, alors même qu’ils sont le résultat du comportement irresponsable de conducteurs qui, délibérément, ont décidé de faire reposer sur autrui le poids de leur insouciance fautive. Il était donc urgent de répondre au sentiment des victimes et de leur famille, que l’emploi de l’adjectif « involontaire » pouvait heurter en venant leur infliger une forme de double peine. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale faisait écho au combat mené par les associations de victimes. J’ai pour elles une pensée compatissante, et je tiens surtout à leur témoigner ma reconnaissance pour leur engagement. Conformément aux recommandations du comité interministériel de la sécurité routière, l’objectif principal est de faire la distinction entre un « homicide volontaire » et un homicide qualifié de « routier », selon l’existence, ou non, de circonstances aggravantes. Sans circonstance aggravante, c’est la qualification d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire qui sera retenue, tandis que, en présence d’une ou de plusieurs circonstances aggravantes, ce sera celle d’homicide routier et de blessures routières. Cette Cette évolution sémantique répond à une attente forte et légitime. En effet, si pour les juristes la qualification d’homicide involontaire peut faire sens, elle perd toute pertinence et se révèle même insultante pour les victimes et leur famille lorsque c’est tout à fait sciemment que des conducteurs prennent le volant sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants. En plus de cette modification importante, le texte initial comportait l’ajout de circonstances aggravantes permettant de qualifier l’homicide routier ou les blessures routières. Ces deux nouvelles qualifications étaient susceptibles d’une condamnation aux mêmes peines complémentaires que pour les homicides ou atteintes involontaires. Certaines d’entre elles voyaient toutefois leur champ d’application et leur durée élargie. Je tiens à saluer le travail des députés, plus particulièrement celui de la rapporteur, Mme Anne Brugnera, dont les travaux ont permis l’adoption de dispositions visant précisément à mieux lutter contre les comportements dangereux au volant et à renforcer la répression à l’égard des auteurs d’infractions routières. Ainsi, les excès de vitesse de 50 kilomètres par heure et plus sont constitutifs de délits ! les règles en matière de récidive ont été renforcées et la suspension administrative du permis de conduire devient systématique à l’encontre d’un conducteur sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool. Si la commission des lois au Sénat souscrit à la volonté de créer un homicide routier, elle a toutefois souhaité aller au delà du dispositif initial proposé par l’Assemblée nationale. l’initiative de son rapporteur, notre collègue Francis Szpiner, dont je salue le travail, elle a fait le choix de systématiser la nouvelle qualification d’homicide routier à tous les homicides ou blessures commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, que le conducteur ait eu un comportement à risque ou non. Cette rédaction de l’article 1 conduit à faire disparaître les infractions « involontaires » pour les accidents de la route, même en cas de simple maladresse ou d’imprudence. Or le groupe RDPI estime que c’est justement cette distinction entre l’homicide involontaire et l’homicide routier qui fait la pertinence de ce texte, car elle met efficacement la lumière sur les situations où le conducteur a délibérément aggravé le risque d’accident. Nous soutiendrons donc en séance un amendement dont les dispositions vont dans le sens du rétablissement de la rédaction initiale. Autre modification apportée en commission au Sénat, l’instauration d’une peine plancher pour les homicides routiers par mise en danger. Ici encore, nous comprenons la volonté de renforcer la lutte contre les violences routières et de mieux sanctionner les comportements fautifs et à risque. Toutefois, nous craignons que, par cette mesure, nous n’ouvrions un débat autour du sujet sensible des peines planchers, débat qui serait,, préjudiciable à l’adoption effective du texte. Nous n’imaginons pas une seconde que cela puisse être le souhait de M. le rapporteur, tant le sujet des violences routières et la lutte contre ce fléau sont des questions qui nous rassemblent tous bien au delà de nos appartenances politiques. Sur le fond, s’il est vrai que le juge, en l’espèce, garde une marge de manœuvre, puisqu’il conserve la faculté de déroger au prononcé d’une peine plancher, il ne peut le faire qu’à condition de motiver spécialement sa décision.

En conclusion, nous notons que l’objectif de ce texte fait largement consensus dans les rangs de notre assemblée et que nous avons tous à cœur de mieux lutter contre les violences routières. Nous craignons toutefois que le mieux puisse être l’ennemi du bien. Aussi nous inscrivons nous en faux par rapport à certaines positions de la commission, qui risquent de compliquer le parcours législatif du texte. Nous en appelons à la responsabilité de chacun,

nous savons que, en 2023, 3 400 personnes sont décédées dans un accident de voiture, de moto ou de mobylette. Tout ce qui peut être fait pour lutter contre ces drames doit être fait.

pour les familles qui ont perdu un proche. C’est le cas de la famille du jeune Antoine Alléno, tué par un

tout accident mortel comme étant un homicide routier, dès lors que la personne n’était incontestablement pas en situation de conduire son véhicule. C’est là que réside l’écart avec la proposition de M. le rapporteur,

qui est bien de stigmatiser et de punir de manière plus forte ceux qui ont conduit dans un état ne le permettant pas. Vous introduisez une confusion juridique en créant une troisième sorte d’infraction

la double peine : voilà ce que ressentent les familles endeuillées lorsque le chauffard qui a mortellement percuté un être qui leur est cher n’effectue aucun jour d’enfermement. Ce n’est pas un cas exceptionnel. C’est plutôt courant, et cela même quand le meurtrier a 2 grammes d’alcool dans le sang. C’est l’histoire qu’a vécue Guillaume, 21 ans, mortellement fauché, en 2017, à Amiens. Une triste réalité à laquelle ont été confrontés mes collègues sénateurs de la Somme, Laurent Somon et Stéphane Demilly, avec lesquels j’avais déposé une proposition de loi, afin que plus aucune famille n’ait à subir cette humiliation,

bien avant l’affaire médiatique d’un célèbre humoriste français, qui a poussé le Gouvernement à réellement traiter la question des violences routières. Nos travaux visaient à améliorer l’effectivité des peines.

Ce texte est ainsi l’occasion de mettre fin au mépris de ces délinquants routiers qui passent entre les mailles d’un filet juridique fragile et totalement inadapté à la réalité de ces drames. d’« homicide involontaire » est insupportable. C’est pourquoi je soutiens pleinement la création d’un délit d’« homicide routier », votée à l’Assemblée nationale. Ce changement sémantique est un premier pas attendu par les familles des victimes. regret, le texte initial ne comportait rien sur l’effectivité des peines prononcées. En 2022, sur 192 personnes condamnées pour homicide routier sous l’empire d’alcool ou de stupéfiants, seules 7 ont été placées en détention à la suite de l’audience. Ce sont les chiffres du ministère de la justice. de notre réponse, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce doit être une plus grande fermeté dans l’application des peines et une meilleure prise en charge des victimes. Comment est il encore possible que les victimes ne soient pas tenues au courant de la date de l’audience, ce qui leur permettrait de décider si elles prendront la parole pendant les débats ? Comment expliquer que les parties civiles ne sont pas informées des modalités d’exécution

nous faut donc, ensemble, parfaire ce texte et nous montrer à la hauteur. Pour Noé, pour Antoine, pour Guillaume, pour leurs familles et pour toutes les victimes de comportements intolérables et d’actes meurtriers sur les routes, les sénateurs du groupe Les Républicains répondront présents.

la voiture est essentielle à la mobilité de nos concitoyens dans bon nombre de nos territoires, mais on doit pouvoir se déplacer sans risquer sa vie. Chaque année, 3 000 Français meurent sur la route. C’est inacceptable Les causes des accidents sont multiples : la fatigue, de mauvaises conditions météorologiques, ou encore une faible visibilité. L’État réalise de nombreux contrôles pour assurer la sécurité des automobilistes.

la voiture ne doit pas devenir un bureau ambulant. Malgré les contrôles, malgré les radars automatiques, malgré les actions de prévention, certains de nos concitoyens continuent d’adopter des comportements dangereux, qui ont trop souvent des conséquences tragiques.

Au delà de l’alourdissement des sanctions, le texte vise à distinguer de l’homicide involontaire celui qui est commis sur la route dans des circonstances d’imprudence d’une particulière gravité. Il est en effet incompréhensible, pour les familles de victimes, d’entendre parler d’homicide involontaire lorsque celui qui a tué avait pris le volant en étant ivre ou drogué. En commission, le rapporteur a constaté que les circonstances particulièrement graves dans lesquelles l’homicide est commis ne permettent pas d’alourdir encore les peines encourues, sauf à faire de cette infraction un crime.

Sans être particulièrement partisans des peines planchers, nous n’y sommes pas opposés. Il ne nous semble cependant pas opportun de réintroduire dans notre droit ce dispositif à l’occasion de cette proposition de loi. Le texte vise en outre à renforcer la répression d’une multitude de délits routiers. Il élargit la notion de récidive afin de sanctionner plus sévèrement les auteurs réguliers d’infractions routières. Les excès de vitesse figurent parmi les infractions les plus fréquentes. Ils sont responsables de plus d’un quart des morts sur les routes. Il est envisagé, dans cette proposition de loi, de punir les excès de vitesse supérieurs à 50 kilomètres par heure non plus comme des contraventions, mais comme des délits. Notre groupe ne peut que soutenir cette disposition. Nous soutenons également le renforcement des sanctions encourues par les automobilistes qui prennent le volant en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants. L’actualité fait trop souvent état d’accidents mortels commis par des individus suffisamment irresponsables pour prendre le volant après avoir consommé de l’alcool ou des drogues, qui ensemble sont responsables de 41 % de la mortalité sur la route. Il est urgent d’y remédier. Le texte alourdit les peines encourues pour la conduite sous l’effet de l’alcool ou de drogues. Il aggrave encore les peines encourues par ceux qui cumulent ces deux états. Nos concitoyens attendent en la matière la plus stricte fermeté. Pour renforcer encore l’effet de ces sanctions, le texte prévoit de rendre systématiques l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule conduit en état d’ivresse ou sous l’empire Nous ne devons négliger aucun moyen pour améliorer la sécurité de nos routes. La proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer contient des dispositions intéressantes, allant vers plus de fermeté.

En 2022, 3 550 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Près de 25 % d’entre elles ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sous la double influence de l’alcool et de stupéfiants. En 2023, 232 000 personnes ont été blessées en France métropolitaine ; 16 000 d’entre elles, grièvement. Face à ces chiffres dramatiques, nos collègues députés ont entendu répondre aux préconisations de portée législative du comité interministériel de la sécurité routière. Sa dixième recommandation était de « créer une qualification d’homicide routier » destinée à « renforcer la valeur symbolique de l’infraction d’homicide dit involontaire ». L’objectif est de « permettre une meilleure acceptation sociale d’une telle qualification ». Comment Comment des parents, en effet, peuvent ils entendre que l’accident qui a causé la mort de leur enfant est involontaire, lorsque le conducteur qui l’a provoqué a pris le volant ivre ou sous l’influence de drogues, ou lorsqu’il roulait plus de 30 kilomètres par heure au delà de la vitesse autorisée ? C’est inaudible, c’est inacceptable Permettez moi de saluer les travaux antérieurs de certains de nos collègues dans le domaine plus large de la sécurité routière, que ce texte laisse sur leur faim.

une ou plusieurs circonstances aggravantes. Nous devons reconnaître le caractère délibéré des violences routières. Celui qui boit sait qu’il boit. Celui qui se drogue sait qu’il se drogue. Celui qui roule trop vite sait qu’il roule trop vite. C’est pourquoi je salue la création des infractions d’homicide routier et de blessures routières. Si l’objet de ce texte n’est pas de dénaturer le caractère involontaire de ces infractions au sens juridique du terme, nous devons tenir compte de la réalité : il est insupportable pour les victimes de devoir accepter de façon inconditionnelle l’adjectif « involontaire ». Le texte reprend donc la distinction entre l’homicide routier et les blessures routières

Pour rappel, le tabac est considéré comme une substance psychoactive, au même titre qu’un grand nombre de médicaments utilisés au quotidien. Par ailleurs, nous nous félicitons de l’assimilation de la récidive de plusieurs infractions à un état alcoolique ou à l’usage de stupéfiants. Celui qui, malgré les restrictions apportées à son droit de conduire, prend le volant régulièrement et défie ainsi l’autorité de l’État doit être puni.

l’impérieuse obligation de requérir afin que soient réprimées énergiquement et rapidement les infractions les plus graves, telles que la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, la violation des signaux d’arrêt impératif ou l’excès de vitesse manifeste. Cette politique judiciaire sera poursuivie avec fermeté. étaient les mots qu’en avril 1985 Robert Badinter, dont nous saluons tous ici le parcours politique et la finesse de l’analyse juridique, employait pour évoquer les irresponsables au volant, qui tuent et blessent sur nos routes.

résultant de « réponses législatives à des événements particuliers ». Avec la rédaction actuelle, comment poursuivre une personne ayant volontairement conduit son véhicule dans l’intention préméditée de donner la mort ? La notion de discernement est elle un concept définitivement révolu ?

Mais les actions concrètes de prévention routière sont les grandes absentes de ce texte. « Mais au delà de ces chiffres – est il besoin de le rappeler devant la Haute Assemblée ? – il y a – ce qui est plus important encore – la souffrance des femmes et des hommes meurtris dans leur corps, la douleur et l’angoisse des proches, des époux, des parents, des enfants.

Aucune loi ne pourra, hélas ! les ramener à la vie ou apaiser la douleur de ceux qui restent. Nous sommes sans doute nombreux à connaître, dans notre entourage, une personne qui a perdu la vie dans un accident de la route. Et pour cause : en 2022, 3 550 personnes ont perdu la vie sur les routes en France – ces chiffres sont en hausse. Dans mon département de Meurthe et Moselle, il y a eu 601

sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour un homicide, cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende pour une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne

ce mécanisme contraire au principe constitutionnel de l’individualisation des peines. Sans étude d’impact et sans analyse complémentaire,

de la prévention et de la sécurité routière n’est plus à démontrer. Elle a permis, depuis les années 1970, de faire chuter le nombre de morts sur les routes. Alors pourquoi est elle la grande oubliée de cette proposition de loi ? Nous avions déposé un amendement visant à développer la prévention dès l’âge de 16 ans, lors de la Journée défense et citoyenneté (JDC). Il a été déclaré irrecevable, c’est dommage. De plus, le texte ne contient pas un mot sur la lutte contre la consommation d’alcool au volant, qui est pourtant responsable de 30 % des accidents de la route et des drames qui en découlent. Nous avions également déposé un amendement sur ce point. Il a, lui aussi, a été déclaré irrecevable. Il apparaît donc à lutter contre la violence routière, se cantonne pourtant à un alourdissement des sanctions, sans volet de prévention. Malgré ces regrets, nous ne nous opposerons pas à ce texte, puisque nous souhaitons renforcer la lutte contre la violence routière. Il sera pourtant nécessaire de prendre des mesures préventives pour protéger nos vies et celles de nos proches sur les routes, en sensibilisant chacun, dès le plus jeune âge, aux dangers de la vitesse et de la consommation d’alcool et de stupéfiants et en lançant des campagnes de prévention importantes, sur tout le territoire, afin de toucher tous les conducteurs. Mais il nous faudra aussi nous interroger sur l’opportunité de construire et de vendre des voitures toujours plus puissantes et plus rapides alors que la vitesse, limitée en droit sur nos routes, est la première cause

le texte que nous étudions affecte un grand nombre de nos concitoyens. La mort tragique d’une personne dans un accident impliquant un véhicule ne saurait plus être réduite à un fait divers. Nous savons – les statistiques le confirment – que trois facteurs augmentent particulièrement le risque d’accident : la vitesse, l’alcool et les stupéfiants. trois éléments sont d’ores et déjà réprimés par notre droit pénal, puisqu’ils constituent des infractions en propre, mais également des circonstances aggravantes dans la caractérisation des infractions d’homicide et d’atteinte à l’intégrité physique de la personne. Il nous est ici proposé de créer de nouvelles infractions routières pour éviter que celles ci puissent être qualifiées d’involontaires. Tant pour les auteurs de la proposition de loi que pour le comité interministériel de la sécurité routière, la principale mesure proposée est symbolique.

En effet, notre société ne supporte plus qu’un chauffard qui s’est lui même placé dans une situation qui augmente dramatiquement les risques pour autrui soit condamné pour une atteinte ou un homicide dits « involontaires C’est bien dans cet esprit que le texte a été adopté, à l’unanimité, par l’Assemblée nationale. Lorsque nous créons de nouvelles qualifications pénales, nous devons nous prémunir de deux effets pernicieux. il faut bien se garder de rendre floues les frontières établies, en l’espèce, entre l’intentionnalité et la non intentionnalité de l’atteinte aux personnes. D’autre part, ne perdons pas de vue que la fonction première du droit pénal est de réparer les dommages causés à la société et de sanctionner les atteintes inacceptables. Au regard de cela, le texte adopté par l’Assemblée nous semblait opérer une juste conciliation entre la nécessité de moderniser le droit pénal, notamment pour mieux répondre aux attentes des victimes, et la préservation de ses grands principes. proposition de loi conservait, dans une certaine mesure, un caractère supplétif à l’infraction d’homicide routier, pour sanctionner d’abord la faute intentionnelle qui a pu conduire à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. Elle répondait aux attentes des victimes, sans entrer dans une dérive. Hélas ! le texte adopté par notre commission des lois ne donne pas le même sentiment. Notre Notre rapporteur, dont il faut souligner le sérieux et la qualité des travaux, a proposé d’élargir le dispositif à tous les homicides commis lors d’un accident routier, avec ou sans circonstance aggravante.

Chacun le sait, les peines planchers vont à l’encontre de principes fondamentaux qui guident le droit pénal français. C’est notamment le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation de la peine qui est en jeu.

du RDSE, en accord avec leurs principes, détermineront leur position une fois achevé l’examen des amendements.

la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière. Cette promesse est celle que j’ai faite à Yann Desjardins, dont le fils Guillaume a été fauché en septembre 2017 par un chauffard alcoolisé alors qu’il circulait à vélo.

Il souhaitait que le chauffard à l’origine de la mort de son fils, condamné à porter un bracelet électronique, aille véritablement derrière les barreaux. Il remuait ciel et terre pour cette cause. Cette promesse est celle que j’ai faite à Thibaut, le frère de Guillaume, qui poursuit ce combat pour que la justice entende le besoin d’une qualification d’homicide routier débarrassée de l’insupportable adjectif « involontaire

de graves blessures. Monsieur le garde des sceaux, vous avez affirmé devant l’Assemblée nationale : « En droit, les mots consacrés par la loi ont encore plus de poids, surtout quand il s’agit de qualifier des actes qui ont causé la perte d’un être cher. »

responsable et humaine, à apaiser les douleurs et à convaincre du rôle éducatif et préventif des sanctions et des mesures de prévention. J’ai fait un rêve et une promesse : plus de sécurité routière, moins d’insécurité pénale

prévue en troisième point de l’ordre du jour de l’après midi du mardi 2 avril prochain, soit reportée au mercredi 3 avril à seize heures trente, après les questions d’actualité au Gouvernement.

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi

à tirer les conséquences de la création de l’homicide routier, nouvelle qualification des homicides involontaires résultant d’un accident de la route en présence de certaines circonstances aggravantes.

Mme Corinne Bourcier. Par un décret en date du 20 décembre 2023, le Gouvernement a souhaité abaisser à 17 ans l’âge à partir duquel il sera possible de passer le permis de conduire. Cette mesure, mise en œuvre par voie réglementaire, modifie l’article R. 221 5 du code de la route, qui dispose que les personnes qui souhaitent obtenir le permis B doivent être âgées d’au moins 18 ans. S’il est maintenant possible d’obtenir le permis de conduire plus jeune, il convient d’assumer toutes les responsabilités qui peuvent en découler. Aussi convient il, dans cette proposition de loi, d’abaisser l’âge de la majorité pénale pour les violences routières, afin que ces jeunes conducteurs soient punis comme les adultes.

ces années d’attente épuisent. Pire, elles font naître ou renforcent la méfiance envers l’institution judiciaire. Vous l’aurez compris, cet amendement vise à raccourcir ces délais dans le seul objectif d’assurer une réponse pénale plus rapide aux délits routiers.

Je défends donc un amendement de bon sens, une mesure très attendue par les familles des victimes. Nous proposons que, en l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile soit avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. Les victimes ou leurs proches pourront ainsi demander à prendre la parole, même en l’absence d’appel sur les intérêts civils.

peines par le juge demeure la manière la plus convaincante – si ce n’est la seule – de rendre la justice pénale dans un État de droit.

de prévoir une prise en charge spécifique des principaux facteurs d’accidents routiers dans le cadre de l’accompagnement vers la réinsertion des personnes détenues condamnées pour ce type d’infractions.

Sol. L’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière contraint la personne condamnée à prendre pleinement conscience de la dangerosité de son comportement

Afin de ne pas entraver l’appréciation du juge, il est cependant prévu que celui ci puisse y déroger, mais il devra motiver spécialement sa décision. Cela aura pour vertu de permettre aux parties civiles de mieux comprendre le verdict, et ainsi de lutter contre le sentiment d’injustice trop souvent souligné par les victimes et leurs proches. Reconnaître l’homicide routier, c’est bien ; prévenir les comportements pour éviter qu’ils ne surviennent, c’est mieux. Tel est l’objet de cet amendement.

des comportements d’un grand nombre de conducteurs, particuliers comme professionnels, vers une conduite apaisée et plus respectueuse des règles du code de la route. C’est dans cet esprit que ce code rend le stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximum de points, trois, et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223 1 du même code. Étendre cette mesure à tous les conducteurs qui auraient perdu la moitié de leurs points, en substituant le stage l’amende correspondante, constituerait, de notre point de vue, un mauvais signal, dans la mesure où cela préserverait le droit à conduire et les finances des conducteurs les plus «

et à apprécier l’opportunité de le faire. Elles présentent donc un fort risque de discrimination et de rupture du principe d’égalité devant la justice, ainsi que de rupture d’équité entre les justiciables dans la constatation et la poursuite des infractions pénales. Le Gouvernement ne doit pas oublier

Le recours n’est pas suspensif et les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe s’oppose à l’application de l’AFD aux délits routiers.

Cet amendement vise donc à éviter que certains individus ne continuent à conduire dans l’attente de la décision de justice, en rendant obligatoire la réalisation d’un examen médical permettant d’évaluer l’aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident.

puis scrutin public solennel sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle Calédonie (texte